Monsieur le président, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs,

Ce sont des considérations d'efficacité opérationnelle, de pragmatisme, de respect de l'équilibre initial et de recherche du plus large consensus qui continuent à nous animer collectivement. Je souhaite, à cet égard, remercier particulièrement, au nom du Gouvernement, les membres de la commission des lois du Sénat, mais aussi ceux de la délégation parlementaire au renseignement (DPR) et de la mission d'information sur l'évaluation de la loi Renseignement,

voudrais également saluer nos services de renseignement, nos policiers, nos gendarmes, qui, chaque jour, font un travail exceptionnel pour identifier les menaces, suivre les individus dangereux et mettre en péril leurs projets meurtriers. nouvelle lecture donc, après l'échec de la commission mixte paritaire (CMP). Alors même qu'un consensus, dont nous devons tous nous féliciter, s'est dégagé sur la majorité des dispositions de ce texte relatif à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement, une divergence de vues sur le dispositif de suivi des sortants de prison condamnés pour terrorisme a conduit à cet échec, que nous assumons. Vous le savez, 188 condamnés terroristes islamistes sortiront de détention d'ici à 2025, dont beaucoup demeurent ancrés dans une idéologie radicale. Ces individus, qui constituent le « haut du spectre » des objectifs suivis par les services de renseignement, présentent des enjeux sécuritaires multiples à la sortie de la détention : prosélytisme, menace à court terme, représentée par certains profils impulsifs, menace à moyen et long terme relative à des projets d'attentats ou encore tentatives de redéploiement vers des zones de djihad à l'étranger. L'expérience acquise au cours des dernières années nous permet aujourd'hui d'affirmer que le placement sous Micas (mesures un outil particulièrement utile et adapté : il permet de faciliter la surveillance d'individus sortant de prison, d'observer leurs relations habituelles, leur pratique, leur activité sur les réseaux sociaux, leurs efforts de réinsertion, etc., quand la mise en place d'une surveillance physique ou technique

D'ores et déjà, un certain nombre de Micas- dix-neuf depuis 2017 -sont arrivées à échéance, alors même que les services sont en mesure de justifier de la persistance de la menace constituée par le comportement des individus C'est pourquoi le projet du Gouvernement, voté par l'Assemblée nationale, prévoit, dans des conditions strictement encadrées, un allongement de ces Micas à une durée de deux ans. Je rappelle que cet allongement est accompagné de garanties fortes, qui permettent de sécuriser la mesure sur le plan constitutionnel. Ainsi, la Micas ne pourra être prolongée jusqu'à vingt-quatre mois qu'à l'encontre d'individus condamnés pour des faits de terrorisme à au moins cinq ans de détention, ou trois ans en cas de récidive. En outre, au-delà de douze mois, le renouvellement de la mesure sera soumis à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. En 2018, le Conseil constitutionnel a, il est vrai, fait de la limitation à douze mois l'un des éléments du bilan de la constitutionnalité des Micas. Il s'est cependant prononcé sur une population différente et bien plus large qui est visée par l'amendement du Gouvernement : étaient ainsi concernées, de manière générale, les personnes présentant des signes avérés de radicalisation, y compris celles qui ne sont pas passées à l'acte et qui n'ont donc pas pu faire l'objet d'une judiciarisation. Il s'agit donc de cas différents. En revanche, le juge constitutionnel n'a pas été saisi du cas spécifique du cas spécifique des individus ayant fait l'objet d'une condamnation pour des faits de terrorisme, qui présentent une différence objective de situation pouvant justifier des mesures

depuis 2017 ne serait pas possible sans le soutien constant du Parlement : renforcement des moyens humains, budgétaires et aussi- surtout, oserais-je dire ici -juridiques, au profit de l'ensemble des services de renseignement, des forces de sécurité, des magistrats de l'ensemble des services de l'État qui mènent ce difficile combat sans relâche. La parole

que les moyens pour y parvenir sont multiples. Après l'échec de la commission mixte paritaire, le 9 juillet 2021, l'Assemblée nationale a achevé, le 13 juillet, l'examen en nouvelle lecture de ce projet de loi.

Cette intransigeance s'est confirmée en nouvelle lecture, alors que les points de vue s'étaient fortement rapprochés entre députés et sénateurs juste avant la CMP. Je rappelle que notre principal point de désaccord porte sur les modalités de suivi des personnes condamnées pour des actes de terrorisme sortant de détention. Nous sommes d'accord sur le constat

Le Gouvernement et l'Assemblée nationale proposent d'allonger la durée des Micas à deux ans, afin d'assurer la surveillance de ce public, tout en instaurant une mesure judiciaire qui se concentrerait sur leur réinsertion. de remettre la loi votée en juillet dernier sur le métier, en instaurant une mesure judiciaire à visée non pas seulement de réadaptation sociale, mais également de surveillance de l'individu.

prononcées par un juge, elles offrent des possibilités de surveillance plus longue et potentiellement plus contraignante ; elles présentent des garanties plus importantes pour les individus concernés, car elles sont prononcées à l'issue d'une procédure contradictoire ; elles permettent, enfin, d'associer aux mesures de surveillance des mesures sociales visant à favoriser la réinsertion de la personne. L'Assemblée nationale n'a pas souhaité donner suite à nos multiples propositions de compromis sur l'article 5. Je rappelle que nous en avons pourtant fait douze et que nous avions beaucoup travaillé. Face à cette position intransigeante de la majorité gouvernementale, nous vous proposerons de supprimer les prolongations des Micas à l'article 3, mais d'adopter, à l'article 5, une rédaction qui avait été discutée avec les députés préalablement à la CMP. Il s'agit, afin d'assurer la bonne articulation entre mesure judiciaire et mesure administrative, de prévoir que, lorsque la mesure de sûreté comprend des obligations qui sont similaires à celles prononcées dans le cadre des Micas, les premières ne peuvent entrer en vigueur que lorsque les secondes sont levées. Nous vous proposerons également de rétablir le texte du Sénat à l'article 2. Notre texte permet une caractérisation plus précise des locaux annexes au lieu de culte qu'il sera possible de fermer s'il existe des raisons sérieuses de penser que ceux-ci seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de la mesure de fermeture du lieu de culte. Dans une perspective de conciliation avec l'Assemblée nationale, nous vous proposerons de supprimer la mention de l'accueil habituel de réunions publiques, étant entendu que les mesures de police administrative ne peuvent concerner des lieux privés,

du Sénat a été de doter les services des moyens adaptés pour faire face à l'évolution, notamment technologique, des pratiques terroristes et criminelles qui menacent la sécurité intérieure de notre pays. Notre travail a été guidé par le respect des libertés constitutionnelles, en nous assurant notamment de la protection de la vie privée, par un réel encadrement législatif doublé de contrôles suffisants. En première lecture, le Sénat avait abouti à un juste équilibre entre liberté et sécurité. Après des discussions très constructives avec mon homologue, le député Loïc Kervran, et grâce aux nombreux échanges menés au sein de la DPR, nous étions parvenus à nous entendre sur la partie relative au renseignement. Cet accord n'a malheureusement pas survécu à l'échec de la CMP. Les députés ont rétabli l'accès des services du second cercle à l'expérimentation relative à l'interception des données satellitaires, mais cela ne constitue pas pour nous un point de blocage. L'Assemblée nationale a en effet précisé que les services du second cercle concernés seront ceux dont les missions le justifient et seront déterminés « par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Dès lors, les conditions de participation de ces services nous paraissent satisfaisantes et suffisamment précises. En revanche, à l'article 13, les députés ont supprimé le caractère expérimental de l'extension du traitement par l'algorithme des URL, prévu par le Sénat jusqu'au 31 juillet 2025. Or, d'un point de vue tant technique que juridique, cette extension ne nous paraît pas possible sans une expérimentation préalable. Je rappelle que les URL sont des données de nature mixte, qui relèvent à la fois des données de connexion et du contenu des communications et qu'elles font donc légitimement l'objet d'une protection renforcée. La nécessité d'une expérimentation avait été soulignée par la DPR dans son dernier rapport, et je regrette que nous n'ayons pas trouvé d'accord sur ce point. Nous vous proposerons donc de rétablir la version du Sénat à l'article 13. Outre des modifications purement rédactionnelles, les députés sont revenus sur une précision que nous avions introduite à l'article 15 sur la conservation des données de connexion.

Nous souhaitions inscrire dans la loi que les catégories de données conservées par les opérateurs dans le cadre de leur obligation de conservation permanente, c'est-à-dire les données relatives à l'identité, les coordonnées de contact et de paiement, les comptes et les adresses IP, devaient

que le Sénat avait adopté deux amendements rédactionnels sans modifier la teneur de l'article 7 portant sur la communication d'informations aux services de renseignement par les autorités administratives,

doit néanmoins se faire conformément à nos valeurs. Si nous en changions, nous offririons la victoire aux terroristes. C'est la raison pour laquelle, depuis le début, le groupe socialiste considère que la prévention relève du pouvoir administratif, mais que, dès que c'est possible,

non pas sur des mythes, mais sur la réalité, et de donner la possibilité à nos chercheurs de construire notre récit national sur les faits est essentiel.

En effet, les membres de la commission mixte paritaire n'ont pas divergé sur le principe selon lequel ces sortants de prison condamnés pour des faits de terrorisme doivent faire l'objet d'un suivi, mais plutôt sur la nature et le contenu de ces mesures.

253 sont condamnées et purgent une peine ; 162 devraient être libérées dans les quatre prochaines années et risquent réellement de réitérer leurs actes. Ce risque, nous le savons tous, n'est pas théorique, ces chiffres ne sont pas équivoques : il faut donc agir vite pour mieux protéger nos concitoyens. La question des sortants de prison illustre de façon emblématique l'évolution d'une menace de plus en plus endogène. Aussi, il est de notre devoir de tout mettre en oeuvre pour garantir la protection de nos concitoyens. Ce projet de loi est primordial à bien des égards. Tout d'abord, il touche au droit à la sûreté. Il nous permet de lutter avec plus d'efficacité contre les ennemis de la France, qui veulent nous toucher au coeur. À chaque attaque, c'est la République française tout entière qui est atteinte. Ensuite, ce projet de loi est indispensable à tous ceux dont l'activité, bien souvent dans l'ombre, est de lutter au quotidien contre la menace terroriste. Le terrorisme constitue un défi majeur de notre temps. C'est- il faut le dire -une nouvelle forme de guerre. Chaque jour qui passe nous rappelle à quel point la menace est omniprésente. Elle prend des formes diverses et variées et se nourrit des progrès technologiques. Plus que l'obligation, nous avons le devoir d'y faire face. Nous devons donner aux services de renseignement les moyens de s'adapter à une nouvelle donne à la fois juridique, technologique et opérationnelle. Dans un autre contexte, l'actualité nous le rappelle. Si une menace existe, elle doit être prise en compte. S'il existe un vide juridique, il doit être comblé. Nous avons aussi le devoir d'éviter tout risque constitutionnel. Je pense notamment Je pense notamment à la question de l'allongement de la durée des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. À cet égard, je salue véritablement le travail de la commission des me félicite que le Sénat ait privilégié la voie du renforcement des dispositifs de suivi judiciaire. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte modifié par notre commission. Il fixe le cadre législatif dont nous avons besoin pour améliorer la défense de notre nation contre toutes les formes de terrorisme et, ainsi, garantir la sécurité de nos concitoyens. Comme le disait si justement le général de Gaulle : « La défense ! C'est la première raison d'être de l'État. Il n'y peut manquer sans se détruire lui-même.

ou ne pas vouloir doter les pouvoirs publics des moyens nécessaires pour y faire face. Mais à quel prix ? Au prix de l'affaiblissement des droits et libertés garantis par notre Constitution ? Au prix d'atteintes à la liberté d'aller et venir, au secret des correspondances, au secret professionnel ou encore au droit au respect de la vie privée et familiale Au prix de l'instauration d'une surveillance généralisée de nos concitoyens au moyen d', de captage des données de communication satellitaires et de recueil des URL ? Au prix d'un dessaisissement du juge dans sa mission de protection des libertés individuelles par la pérennisation, dans notre droit commun, du recours intensif à des procédures administratives relevant du cadre de l'état d'urgence ? À quel prix, avions posé la question lors de l'examen de la proposition de loi Justice de proximité et réponse pénale : de quels moyens parlons-nous quand la justice pâtit d'un manque de ressources humaines et matérielles importantes, qui l'empêchent de mener à bien sa mission ?

Et si la seule réponse que souhaite apporter ce gouvernement à la menace djihadiste est d'ordre sécuritaire, il signe dès aujourd'hui l'échec de la politique de prévention des actes terroristes en France.

loi traite par ailleurs de la question des archives : il prévoit de restreindre l'accès à celles-ci- notre collègue Leconte vient d'en parler -, ce qui contrevient à un autre droit consacré au niveau constitutionnel en vertu de l'article XV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

À la place, le choix est arbitrairement fait de s'attaquer aux archives et d'inscrire dans notre droit des procédures exorbitantes du droit commun, qui viennent affaiblir peu à peu notre État de droit. Comme nombre de défenseurs des libertés publiques, nous tirons la sonnette d'alarme : pouvons-nous réellement concevoir une société vivant dans un état d'urgence permanent ? L'accumulation et la pérennisation des lois d'exception- il s'agit là du huitième texte de cette nature depuis 2015 -ne sont jamais de bon augure. Je regrette de surcroît l'absence totale de concertation préalable, tout comme je dénonce le recours à la procédure accélérée dont le Gouvernement a pris l'habitude : tous deux privent le Parlement d'un véritable débat. débat. S'agit-il réellement d'une manoeuvre politicienne consistant à cranter les thématiques régaliennes dans le débat public à l'approche de l'élection présidentielle ? Chacun se fera son opinion sur la question. En ce qui concerne le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, nous ne saurions l'accepter. Comme en première lecture, nous voterons contre ce texte.

des menées terroristes qui continuent à être ourdies dans notre pays. Le présent projet de loi conduit à consolider les outils principaux de surveillance antiterroriste que sont les Micas, les contrôles des lieux de culte, les visites domiciliaires et les périmètres de protection, en leur

même s'il est vrai qu'elle est partielle -au défi légal posé par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la conservation des données, telle que l'a interprétée le Conseil d'État il y a quelques semaines.

et au vu de l'expérience désormais prolongée des services compétents, que la durée de la mesure administrative, même portée à deux ans, est adaptée à la situation et qu'elle peut être sécurisée juridiquement- nous le verrons bien dans quelques semaines. C'est la raison pour laquelle nous défendrons cette formule aux côtés du Gouvernement.

Je le regrette d'autant plus que, sur de nombreux points, nous partons des mêmes constats. Le premier est celui de la nécessité légale. Comme cela a largement été souligné au cours de la navette, à défaut d'une intervention du législateur, bon nombre de dispositions du code de la sécurité intérieure, issues notamment de la loi SILT, arriveront à échéance en 2021. Le second est, bien entendu, l'objet de toutes ces lois : répondre à la menace terroriste et notamment au risque que représente la sortie de détention, dans les prochaines années, de détenus condamnés pour des faits en lien avec le terrorisme. Ce point spécifique doit faire l'objet d'une réponse législative en raison de la particulière dangerosité que présentent ces détenus, pour lesquels le risque de récidive est significativement élevé.

De son côté, l'Assemblée nationale n'a pas changé de position. Elle estime qu'il revient au tribunal de l'application des peines d'ordonner des mesures judiciaires de prévention et de la récidive terroriste et de réinsertion. Ce dispositif aurait pour spécificité de ne contenir que des obligations tendant à la réinsertion des individus concernés, laissant ainsi à d'autres mesures- les Micas prévues à l'article 3, en l'occurrence -le soin d'exercer un contrôle administratif et de surveillance. Notre chambre, quant à elle, prévoyait une mesure de nature administrative, dont le contenu serait mixte : il s'agissait d'un dispositif tant d'accompagnement à la réinsertion que de surveillance, susceptible d'être davantage contraignant. De ce point de vue, donc, la position du Sénat paraissait cohérente et claire dans sa mise en oeuvre. Je crois que l'argument n'était pas qu'accessoire : il compte pour que notre droit fasse preuve de clarté face à l'épreuve que lui impose le terrorisme. notre commission a démontré sa capacité à élaborer un compromis en adoptant, lors de ce nouvel examen, une version remaniée du texte. Elle s'est montrée soucieuse de l'articulation des mesures administratives et de la nouvelle mesure judiciaire qui semblait préoccuper le Gouvernement et l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, la disposition proposée par le Sénat offre des garanties suffisantes au regard du but à atteindre. Surtout, elle ne devrait pas faire l'objet d'une censure de la part du Conseil constitutionnel, ce qui, je le rappelle, est l'une des raisons pour lesquelles nous devons encore nous réunir sur ces questions. En dernier lieu, je veux rappeler notre inquiétude concernant l'article 19 du projet de loi, qui vient définir le régime juridique de la communicabilité applicable aux archives intéressant la défense nationale.

en abordant l'examen en nouvelle lecture d'un texte dont les mesures nous sont désormais, hélas, plus que familières, je dois vous faire part de l'inquiétude doublée d'amertume que nous ressentons au sein de notre groupe, nous qui, comme d'autres,

Ce projet de loi s'inscrit dans la continuité d'une multitude de lois sécuritaires, dérogatoires au droit commun, votées sans véritable évaluation préalable des dispositifs existants, de leur nécessité et de leur efficacité. En votant ce projet de loi, mes chers collègues, vous pérenniserez les dispositifs issus de la loi SILT, c'est-à-dire des dispositifs semblables à des assignations à résidence et à des perquisitions contrôlées par l'administration qui, contournant la procédure judiciaire et les droits de la défense, ont des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes visées, jugées sous couvert d'un motif

vous êtes pourtant d'accord sur la philosophie globale de ce genre de mesures. En réalité, quels que soient l'issue de ce texte et les micro-aménagements sur lesquels vous vous entendrez en pérennisant toutes ces mesures, vous faites le choix d'opérer un tournant radical en matière de police administrative, inspiré par un principe de précaution incompatible avec nos principes démocratiques, fondés sur un droit pénal d'interprétation stricte. Concernant le volet renseignement, ce projet de loi consacre ce qui émergeait déjà dans la loi de juillet 2015 relative au renseignement, qui avait été déférée devant le Conseil constitutionnel par François Hollande lui-même l'extension du champ des activités du renseignement et la légalisation de techniques de surveillance intrusives, en parallèle d'un maintien à distance de l'autorité judiciaire. Avec l'ensemble de ces techniques, le Gouvernement se dote d'un arsenal de surveillance de masse. Pourtant, je vous le redis, nos concitoyennes et concitoyens ne veulent ni renoncer à leur liberté individuelle ni échanger leur vie privée contre un État sécuritaire sans faille, illusoire. Nous nous interrogeons toujours sur l'utilité de ces mesures de durcissement de l'arsenal répressif et administratif antiterroriste, alors même que notre législation en la matière est déjà substantielle.

-n'avait permis d'atteindre aucun objectif opérationnel, et ce alors même que vous ne cessez de nous expliquer que toutes les mesures prises en matière de renseignement sont absolument efficaces et nécessaires pour le travail de nos services de renseignement. Je le redis ici, nous considérons pour notre part que, s'il y a lieu de réformer le renseignement, c'est pour accroître ses personnels et non pour recourir de façon irrationnelle et déraisonnable à des techniques de surveillance massive

la France fait face depuis 2015 à de nombreuses attaques terroristes, certaines d'origine endogène et perpétrées par des personnes se radicalisant sur le territoire national. Outre le risque djihadiste, les services de renseignement s'inquiètent de l'émergence de radicalités multiformes : politiques, religieuses, survivalistes ou encore conspirationnistes.

Le présent projet de loi vise à adapter notre droit à la menace terroriste en apportant une réponse légale et proportionnée aux menaces auxquelles nous continuons de faire face aujourd'hui.

par la loi SILT, comme la fermeture administrative des lieux de culte, des mesures de surveillance ou encore un renforcement des pouvoirs de police administrative. Il crée, de plus, une mesure judiciaire de réinsertion sociale antiterroriste

et a démontré l'utilité opérationnelle pour l'autorité administrative, ainsi que le caractère finalement complémentaire entre l'intervention de l'autorité administrative et celle de l'autorité judiciaire- ce n'était pas forcément acquis initialement.

Nous regrettons bien sûr, comme les collègues qui se sont exprimés avant moi, comme l'a fait également à diverses reprises le président de la commission des lois, que la CMP n'ait pu aboutir sur ce texte. C'est dommage ; l'objectif était à notre sens atteignable.

Or l'Assemblée nationale et, semble-t-il, le Gouvernement n'ont pas souhaité aller au-delà des obligations de réinsertion que nos collègues députés avaient adoptées en première lecture. En réintégrant les articles 3 et 5 dans leur intégralité, articles pourtant modifiés par le Sénat, l'Assemblée nationale a pris la responsabilité de ne pas permettre un accord entre nos deux chambres.

pour lequel la commission a retenu que les incertitudes tant techniques que juridiques liées à l'atteinte aux libertés représentée par la possibilité d'utiliser les URL parmi les données traitées par algorithme

points montre que la rédaction retenue par notre assemblée présentait de nombreux avantages. C'est pourquoi le groupe des sénateurs UC votera en faveur du projet de loi, dans la version issue des travaux de notre commission des lois. La parole est

relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, après l'échec de la commission mixte paritaire du 9 juillet. Cet échec est fort regrettable tant l'accord était atteignable, suite aux discussions constructives entre les rapporteurs de l'Assemblée nationale et nos deux rapporteurs, spécialistes de ces sujets- Agnès Canayer, membre de la délégation parlementaire au renseignement, et Marc-Philippe Daubresse, qui assure le suivi et l'évaluation depuis trois ans de la loi SILT. Comment expliquer cet échec, alors que nous partageons, avec nos collègues députés et le Gouvernement, le constat selon lequel nous ne disposons pas d'outils techniques et juridiques suffisants pour lutter contre le terrorisme ? Ce projet de loi avait vocation à combler ces carences. Je tiens à saluer la position de la commission des lois du Sénat, qui a choisi, non pas de présenter une motion tendant à opposer une question préalable, mais de poursuivre la discussion du texte. En effet, un certain nombre de modifications apportées par le Sénat ont été retenues par la CMP, notamment sur le volet renseignement. Notre collègue rapporteur Agnès Canayer et son homologue à l'Assemblée nationale, Loïc Kervran, étaient parvenus à un accord sur un grand nombre d'articles, afin de donner aux services de renseignement les moyens de lutter contre les nouvelles menaces. Pour cette dernière lecture, notre rapporteur a également accepté les ajustements opérés par l'Assemblée nationale à l'article 7 en matière de communication d'informations aux services de renseignement par les autorités administratives, à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel. l'expérimentation du traitement des URL par l'algorithme, et nous la suivons dans cette voie de prudence. Les rapporteurs ont tenté de trouver un accord, en proposant des solutions acceptables. Il s'avère que leur volonté d'aboutir à un compromis s'est heurtée à l'intransigeance du Gouvernement. Celui-ci ne semble pas apprécier à sa juste valeur l'expertise de la Haute Assemblée et, surtout, sa détermination à apporter de vraies réponses, robustes, efficaces, pour faire face aux menaces qui gangrènent la sécurité de nos concitoyens. Quels sont les principaux sujets qui cristallisent les désaccords entre nos deux assemblées ? Nous les relevons dans le volet relatif à la prévention du terrorisme, domaine ô combien préoccupant. À l'article 2, nous considérons que la formulation retenue par les députés pour définir les lieux annexes aux lieux de culte est insuffisamment précise et comporte un risque constitutionnel qui fragilise le dispositif. En effet, les députés prévoient que ces lieux soient définis comme des locaux dépendants du lieu de culte, alors que nous tenons à préciser qu'il s'agit des locaux gérés, exploités ou financés directement ou indirectement par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte. Nous considérons que la fermeture de ces locaux annexes permettrait de lutter contre le phénomène de déport de certains prédicateurs, qui utilisent ces lieux pour échapper aux mesures de police administrative, ce que soulignait notre rapporteur Marc-Philippe Daubresse dans son rapport d'information sur le suivi de la loi SILT en février 2020. 2020. Notre divergence majeure, à l'origine de l'échec de la CMP, porte sur les articles 3 et 5. Nous l'avions déjà bien perçu lors de la première lecture, madame la ministre, puisque vous aviez déposé des amendements pour rétablir le texte de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas favorables à l'allongement de la durée des Micas. Faut-il rappeler une fois de plus la décision du Conseil constitutionnel, qui a considéré que, compte tenu de leur rigueur, les Micas ne sauraient excéder, de manière continue ou non, une durée totale de douze mois ? J'ai du mal à comprendre pourquoi les députés et le Gouvernement ne comprennent pas cet arbitrage et s'entêtent à vouloir passer cette durée à vingt-quatre mois, et ce malgré les arguments, madame la ministre, que vous avez développés lors de votre intervention en début de séance. Nous soutenons nos rapporteurs, qui ont réintroduit, à l'article 5, la proposition de loi du président Buffet que le Sénat avait adoptée en mai dernier, créant une mesure judiciaire de suivi et de surveillance. Cette dernière semble constituer une voie juridiquement plus adaptée que la proposition initiale du Gouvernement, reprise en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale. Elle offre des possibilités de surveillance plus longue, plus contraignante et permet d'associer aux obligations de surveillance des mesures sociales de réinsertion. Cette mesure reprend le principe du dispositif adopté par le Parlement en juillet 2020, instaurant un régime de sûreté à l'encontre des sortants de prison condamnés pour terrorisme, tout en y apportant les aménagements nécessaires pour répondre aux objections du Conseil constitutionnel. Elle constitue, selon nous, la voie à suivre pour répondre à cette problématique d'une importance toute particulière. Ces dispositions nous paraissent être les plus efficaces et les plus respectueuses des libertés. Tout au long de l'examen de ce projet de loi, nos rapporteurs ont veillé à assurer un équilibre entre les mesures de sécurité et le respect des libertés constitutionnelles. L'enjeu de ce texte est majeur. Il faut renforcer notre arsenal législatif pour assurer la protection de nos concitoyens, qui aspirent à vivre dans un État de droit en toute sécurité. Nous pensons que le texte de l'Assemblée nationale ne répond pas complètement à ces enjeux. C'est pourquoi nous sommes satisfaits que le Sénat imprime sa marque et réaffirme sa volonté de fermeté et d'efficacité, mais aussi d'humanité. Les membres du groupe Les Républicains voteront le texte proposé par nos rapporteurs.

dix. La séance est reprise. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Je mets aux voix l'article 1. bis L'amendement

qu'une personne faisant l'objet d'une telle mesure peut se voir imposer deux séries d'obligations alternatives : d'une part, l'assignation géographique et l'obligation de pointage auprès des services de police ou des unités de gendarmerie ; d'autre part, l'interdiction de paraître dans certains lieux et le signalement de tout déplacement à l'extérieur d'un périmètre défini. Dans les deux cas, le ministre de l'intérieur peut également prononcer une interdiction d'entrer en relation avec une ou plusieurs personnes, ainsi qu'une obligation de déclarer son domicile. La durée des Micas est, à ce jour, strictement encadrée. Comme cela a été dit, ces mesures sont renouvelables uniquement dans la limite d'une durée cumulée de douze mois. Au-delà de six mois, des éléments nouveaux ou complémentaires sont requis pour les prolonger. Prétendant que, pour des profils présentant une dangerosité élevée, la limite de douze mois

un des éléments du bilan de la constitutionnalité de la Micas, il n'a pas été saisi de la différence objective de situation entre les personnes radicalisées n'ayant pas été condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme et celles qui ont fait l'objet d'une condamnation. Pour notre part, nous restons convaincus que, comme l'a exprimé le Conseil constitutionnel dans le commentaire de sa décision, « quelle que soit la gravité de la menace qui la justifie, une telle mesure de police administrative ne peut se prolonger aussi longtemps que dure cette

de paraître ne pouvant être prononcée qu'à l'égard de personnes astreintes aux obligations les plus légères. Or il peut arriver que se tiennent, à l'intérieur du périmètre au sein duquel une personne est astreinte à résider, des événements ponctuels exposés, par leur ampleur ou par leurs circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Je pense, par exemple, à un procès d'auteurs d'actes de terrorisme qui aurait lieu au tribunal judiciaire de Paris, auquel une personne astreinte à résider à Paris pourrait se rendre Actuellement, lorsqu'une telle situation se présente, il est nécessaire de modifier le régime sous lequel est placée la personne pour la placer sous celui de l'article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure, qui permet de prononcer une interdiction de paraître. Dans ce cas, la personne n'est plus astreinte à résider au sein d'un périmètre de résidence et peut le quitter sans encourir aucune poursuite pénale. La mesure proposée dans l'article 3 corrige cette anomalie, en permettant de cumuler l'astreinte à résidence dans un périmètre déterminé et l'interdiction de paraître dans un lieu précis inclus dans ce périmètre et dans lequel se tient un événement particulièrement exposé à raison, soit de son ampleur, soit des circonstances particulières, au risque de menace terroriste.

dont le terme surviendrait moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée supplémentaire de sept jours, s'il est procédé à la notification de leur renouvellement au plus tard le lendemain de la publication de la loi. Cet allongement du délai répond à la nécessité de procéder au renouvellement de nombreuses mesures

est à M. Guy Benarroche. Cet article est celui qui a cristallisé le plus d'oppositions. Il reprend les dispositions de la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine, censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2020. Auparavant, le Conseil d'État s'était déjà interrogé sur l'utilité d'une telle mesure de sûreté. Dans son avis publié le 23 juin 2020, il a énoncé que « la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit permet l'application de presque toutes les mesures de la proposition de loi ».

du code de procédure pénale ou encore le suivi post-libération, prévu à l'article 721-2 du même code. Si nous prenons très au sérieux la nécessité de prévenir la commission d'actes à caractère terroriste, la gravité de ces actes ne dispense pas d'apprécier la stricte nécessité des mesures prévues.

Mme Michelle Gréaume. L'article 6 autorise la communication aux préfets et à certains services de renseignement des données à caractère personnel issues du fichier relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement lorsqu'un patient représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste. Le décret du 6 mai 2019 autorise déjà l'interconnexion du fichier Hopsyweb avec le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste

L'extension du nombre de personnes ayant accès aux informations médicales contrevient aux principes du droit au respect de la vie privée et au secret des informations médicales. Comme l'indique le Syndicat de la magistrature, la lutte antiterroriste, dotée d'un arsenal législatif pléthorique, continue à servir de prétexte à la création de toutes sortes de dispositifs exorbitants, tels que le fichage et le traçage des personnes atteintes de troubles mentaux, sans qu'aucune corrélation ait été établie entre radicalisation à caractère terroriste et troubles psychiatriques

nous considérons que ce débat n'est pas à la hauteur de l'enjeu ; nous y reviendrons lorsque le Gouvernement présentera le projet de loi sur l'irresponsabilité pénale. Pour l'heure, nous vous proposons de supprimer cet article, dont la teneur devrait être éclairée par des travaux divers et pluralistes, encore inexistants. Quel

acte la fin du principe selon lequel les renseignements ne peuvent être utilisés pour des finalités autres que celles qui motivent la procédure de surveillance. En effet, il prévoit la transmission de renseignements entre services et étend par là-même la communication d'informations aux services de renseignement. Autant le dire clairement : cet article est attentatoire aux libertés publiques. En permettant à des services de contourner les restrictions quant à l'usage des dispositifs de surveillance, et en signant la fin du principe de « finalisation », il contrevient au droit au respect de la vie privée. De même, l'absence de contrôle préalable aux mesures de surveillance est problématique. De ce fait, l'article 7 s'inscrit dans la longue liste des dispositions qui poussent à la déjudiciarisation du contrôle en matière de sécurité intérieure.

l'équilibre du texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale et la commission des lois du Sénat, et de concilier le droit à la vie privée et l'efficacité opérationnelle. Seront soumises à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la CNCTR, les transmissions de renseignements « bruts » motivées par une finalité différente de celles qui ont justifié la mesure de surveillance. Il en ira de même des transmissions de renseignements « bruts », transcrits

à tout type d'individu, sans distinctions. La mise en oeuvre de mesures de filtrage en amont pour empêcher toute intrusion serait plus respectueuse de la vie privée des personnes qui ne sont pas visées par la recherche de renseignements. Nous ne sommes pas forcément opposés à l'expérimentation de cette technique dans le seul cadre de la prévention d'actes terroristes. En revanche, votre attention sur le risque d'intrusion trop important, au détriment du droit au respect de la vie privée. Le manque de mesures préventives pour empêcher toute atteinte de ce type est inquiétant. Pourquoi ne pas prendre le temps d'affiner l'expérimentation de ce dispositif,

par être pérennisée. En effet, comme l'indique l'Observatoire des libertés et du numérique (OLN), « il n'y a jamais de retour en arrière sur les expérimentations et mesures liberticides mises en place, aucun retour plus favorable aux libertés », et cela quand bien même des demandes légitimes et mesurées seraient avancées, comme l'augmentation des pouvoirs de la CNCTR, le contrôle des échanges avec des services étrangers, la garantie d'un réel pouvoir de contrôle parlementaire ou la possibilité

Par cet amendement, nous nous opposons à l'extension de la portée des « boîtes noires » au-delà des données de connexion, pour intégrer des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, soit les URL. Je souhaite rappeler notre ferme opposition à la pérennisation des « boîtes noires ». Leur extension est ici orchestrée sans aucun argument précis ni information chiffrée, et sans que soit pris en compte l'avertissement du Conseil d'État.

C'est ignorer la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2015, par laquelle celui-ci avait validé les « boîtes noires », en prenant en compte l'impossibilité qu'elles traitent le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre

est susceptible de faire apparaître des informations relatives au contenu des éléments consultés ou aux correspondances échangées qui ne respecteraient pas la vie privée de la personne- par exemple l'orientation sexuelle, l'état de santé, etc.

En leur qualité de législateur et au regard de leur mission de contrôle de la politique publique du renseignement, les membres de la DPR doivent disposer de ces éléments pour savoir si des contournements au cadre juridique qu'ils ont posé ont été constatés afin, le cas échéant,

qui s'inspire du travail mené sur le sujet à l'Assemblée nationale, tend à modifier la composition de la délégation parlementaire au renseignement et à renforcer ses prérogatives. La DPR n'est actuellement composée que de quatre députés et de quatre sénateurs, dont les présidents des commissions permanentes chargées des affaires de sécurité intérieure et de défense, qui en sont membres de droit. Par le présent amendement, nous souhaitons renforcer son effectif en le portant de huit à vingt membres, afin d'accroître le pluralisme politique de cet organe et de permettre la représentation des groupes minoritaires et d'opposition. Pour gagner en effectivité, la délégation parlementaire au renseignement doit également disposer d'un pouvoir d'injonction renforcé et être en mesure de donner des instructions générales aux services de renseignement. Quel est l'avis de la commission

M. Yannick Vaugrenard. Voilà six ans, le Parlement avait prévu une disposition particulière permettant à la délégation parlementaire au renseignement d'auditionner chaque semestre le Premier ministre sur l'application des dispositions de la loi Renseignement de 2015. En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, considérant qu'elle était obsolète- ce qu'on peut entendre. Néanmoins, il serait utile de la remplacer par une audition annuelle du Premier ministre sur le réexamen périodique de l'état de la menace qui sous-tend le maintien de la conservation généralisée des données de connexion, comme l'exigent, du reste, la Cour de justice de l'Union européenne et le Conseil d'État. En effet, il est important qu'un contrôle parlementaire puisse s'exercer sur le sujet et que l'exécutif motive sa position. À ce titre, il est donc proposé que la DPR, seule instance bicamérale habilitée à connaître d'informations classifiées, puisque ses membres et son secrétariat sont habilités au secret-défense, puisse s'enquérir de l'évolution de la menace à l'occasion d'une audition annuelle du chef du Gouvernement couverte par le secret de la défense nationale.

je tiens à revenir, dans cette explication de vote, sur l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas voter ce texte, et qui porte sur la question des archives,

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

La séance est levée.